La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 23 avril

Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, c'est avec tristesse que nous avons appris la disparition de notre ancien collègue Henri Weber le 26 avril dernier. Cet universitaire s'était passionné pour la politique depuis l'adolescence. Il connut une jeunesse très engagée dans les Jeunesses communistes, puis lors des événements de mai 1968. Il fut aussi cofondateur de la Ligue communiste. En 1986, il rejoignit le parti socialiste, dont il fut longtemps secrétaire national. 1988, Henri Weber devint conseiller technique au cabinet de Laurent Fabius, alors président de l'Assemblée nationale. De 1991 à 1993, il participa comme chargé de mission aux cabinets de Martin Malvy et du président Louis Mermaz, alors ministres chargés des relations avec le Parlement.

Au cours de ses neuf ans de mandat sénatorial, Henri Weber, membre de la commission des affaires culturelles, intervenait régulièrement dans les débats concernant des secteurs qu'il connaissait particulièrement : l'enseignement supérieur, la culture, ou encore la communication et l'audiovisuel.

2004 à 2014. Avec lui disparaît une figure qui a marqué notre vie politique, une personnalité dotée d'un sens de l'humour dont je me souviens personnellement, un intellectuel érudit et passionné par les débats d'idées, qui avait pour devise d'« agir en homme de pensée et penser en homme d'action

exprimer notre sympathie à son épouse Fabienne Servan-Schreiber, à ses enfants, à ses proches, aux membres

Nous avons noté votre grande prudence pour procéder à un déconfinement sous conditions, par étapes et sur-mesure selon les territoires. Nous sommes néanmoins très dubitatifs quant aux modalités et aux moyens mis en oeuvre, et à cet égard vous ne nous avez pas convaincus. Trop d'ambiguïtés demeurent. Même la question de la fourniture de masques à chaque Français, posée depuis des semaines, n'est toujours pas entièrement réglée et le flou relatif à la reprise de l'école inquiète les parents, les enseignants et les maires. Les principes qui guident vos décisions en la matière ne sont d'ailleurs pas clairs et ne semblent être ceux ni de la réussite scolaire ni de l'égalité des chances entre les enfants. Quant à votre réponse à la crise sociale dramatique qui est devant nous, elle n'est pas, à notre avis, à la hauteur de la situation.

Après vous avoir écouté attentivement hier, je veux vous poser deux questions. Quand et comment allez-vous clarifier toutes les zones d'ombre qui persistent encore, en particulier pour l'école ? Allez-vous enfin mettre l'urgence sociale au coeur de votre politique face à cette crise ?

Je l'ai dit hier, je le répète aujourd'hui, et cet état d'esprit ne me quittera pas : nous devons être à la fois prudents et résolus. Prudents, parce que le déconfinement est un processus risqué, et résolus, parce que ne pas déconfiner serait tout aussi risqué. Nous sommes donc condamnés, d'une certaine façon, à avancer prudemment. C'est la raison pour laquelle j'ai indiqué dans mon propos d'hier que je tenais à ce que les opérations de déconfinement s'effectuent progressivement, avec un pas de temps qui permette, avant qu'une nouvelle étape soit franchie, de vérifier que les mesures prises aboutissent à circonscrire l'évolution du virus.

Le deuxième aspect que j'ai évoqué est celui de la différenciation, de la territorialisation des mesures. Celle-ci se justifie par une raison qui me paraît évidente et qui, j'en suis certain, l'est tout autant dans votre esprit. Vous évoquez la question des écoles.

et très bien les écoles de la ville dont j'ai été maire. Dans certaines écoles, les consignes que nous avons données pourront être mises en oeuvre très facilement en raison de la

les maires, les directeurs d'école et les représentants de l'État pourront entamer un dialogue en confiance et trouver les meilleures solutions pour que l'école reprenne. On peut ne pas être d'accord sur la nécessité de cette reprise

Il y aura donc une discussion locale, territoriale, entre les acteurs de terrain, qui conjugueront leurs efforts pour que l'objectif défini dans cette stratégie nationale puisse être atteint. Vous nous dites, monsieur le sénateur, qu'il y a du flou.

Monsieur le sénateur, si vous pensez qu'il existe une autre méthode pour vaincre une épidémie que de faire confiance à ceux qui sont au plus près du terrain

comptes publics. Plus de 20 000 de nos compatriotes ont été emportés par la pandémie de Covid-19. Pour lutter contre le virus et pour éviter qu'il ne fasse davantage de victimes, la Nation a fait bloc. les soignants n'ont pas fléchi. La deuxième ligne a tenu bon. Et la grande majorité de nos concitoyens a scrupuleusement observé les mesures barrières. Cette unité se révèle précieuse dans le combat contre la maladie. Elle le sera tout autant lors du déconfinement. La coopération de toutes les composantes de la société sera essentielle pour assurer la remise en marche de notre pays. Des baisses considérables d'activité de plusieurs administrations ont eu lieu durant le confinement. C'est le cas de la justice, aujourd'hui quasiment à l'arrêt, qui va devoir se mobiliser fortement pour faire face à d'importants retards. Certaines entreprises chargées de service public, comme La Poste, ont également connu des difficultés, péniblement ressenties par les usagers, mais actuellement en voie d'amélioration. Nous avions également eu l'occasion d'alerter le Gouvernement sur la nécessité de poursuivre la délivrance des permis de construire, afin de ne pas mettre en péril la reprise des chantiers le jour du déconfinement. Sur ce point, nous avons été entendus. Cependant, nous continuons d'être sollicités par des entrepreneurs dont l'activité est suspendue du fait de l'absence de décision de l'administration. C'est notamment le cas des chantiers de rénovation énergétique. Les contrôles de qualité, qui doivent être relancés par l'administration pour permettre le financement de ces chantiers les certificats d'économies d'énergie (CEE), sont à l'arrêt. Ce blocage, bien réel, n'est qu'un exemple parmi d'autres qui risquent d'entraver le redémarrage de notre économie. Les entreprises ont besoin de visibilité et de flexibilité. nous dire quelles mesures le Gouvernement a prévu de prendre pour s'assurer que la reprise de l'activité administrative pourra accompagner celle de nos concitoyens ?

vous avez indiqué que certaines administrations avaient dû ralentir leur activité pendant la période de confinement. C'est en effet la réalité, du fait de la mise en oeuvre des plans de continuité d'activité. Au-delà des difficultés que vous avez évoquées et auxquelles nous avons apporté des réponses, souvent par voie d'ordonnance, je veux avant tout retenir le formidable engagement, durant cette période, des agents des trois versants

pour de nombreuses activités économiques, certes assorti de conditions qui méritent d'être précisées, l'horizon d'un retour à une situation normale s'est éloigné pour les festivals, les salles de concert, les théâtres et les cinémas. Il en est de même pour les restaurants, les cafés, les hôtels, les campings, les parcs d'attractions et les voyagistes. L'avenir pour eux reste très incertain.

préféré maintenir un simple report de charges et annoncé des discussions avec les différentes parties. Après vos propos d'hier, je ne doute pas que, face au drame qui s'annonce, vous finirez par suivre le Sénat.

nous devrons continuer d'accompagner ces acteurs. C'est pourquoi nous préparons un certain nombre de mesures d'accompagnement, de soutien et de relance qui seront présentées lors du comité interministériel du tourisme auquel vous participez. Il se tiendra sous la houlette du Premier ministre le 14 mai prochain.

Madame la garde des sceaux, à la suite des annonces que le Premier ministre a faites hier à l'Assemblée nationale, on ne peut que se féliciter de la confiance que le Gouvernement accorde aux territoires pour mener au mieux le déconfinement.

Il reste néanmoins beaucoup de points en suspens. Je pense particulièrement à la responsabilité personnelle, y compris pénale, des employeurs dans le cadre du déconfinement. Alors que le travail doit reprendre, tous se mobilisent : les employeurs du secteur privé, notamment de PME, les employeurs associatifs, mais aussi les employeurs du secteur public, en particulier les collectivités territoriales et les maires. Tous s'organisent de leur mieux pour permettre à leur personnel de réintégrer leur poste dans le strict respect des consignes sanitaires que le Gouvernement a établies et avec les moyens matériels dont ils disposent. Toutefois, le risque zéro n'existe pas.

Je note également les problématiques du respect des règles sanitaires parmi les gens du voyage et de leur installation dans les zones d'accueil. Face aux inquiétudes persistantes, envisagez-vous un éventuel aménagement des règles de responsabilité, hors les cas de faute grave, dans un contexte d'état d'urgence sanitaire prolongé ?

Il serait en effet inconcevable qu'élus locaux, entrepreneurs et employeurs privés s'engagent pour la reprise de l'activité avec la crainte de voir leur responsabilité juridique engagée. Sur ce point, je souhaite vous rassurer. Les règles posées par le code pénal pour engager la responsabilité des élus locaux ou des employeurs privés pour mise en danger de la vie d'autrui ou pour homicides ou blessures involontaires sont restrictives. restrictives. Elles reposent sur la recherche d'un comportement sciemment dangereux, de la prise délibérée d'un risque au mépris de la sécurité des autres. La responsabilité pénale ne peut donc être engagée qu'en cas de

En matière de droit du travail, c'est-à-dire de responsabilité civile, l'assemblée plénière de la Cour de cassation juge que l'employeur qui prend les mesures de prévention nécessaires respecte ses obligations légales en matière de protection de la santé de ses salariés. Autrement dit, l'obligation de l'employeur est une obligation non pas de résultat, mais de moyens renforcés. Au regard de ce cadre juridique, ce cadre juridique, je ne vois pas comment les élus locaux ou les employeurs qui donneraient les instructions nécessaires afin d'assurer le le respect des gestes barrières et des dispositifs de sécurité pourraient voir leur responsabilité engagée. Si des clarifications textuelles apparaissaient nécessaires, nous pourrions évidemment y réfléchir avec vous.

le protocole sanitaire applicable, qui sera publié vendredi, comportera-t-il des préconisations- à mes yeux nécessaires -pour les activités périscolaires, par exemple pour le nettoyage des salles, la restauration et les activités de garderie ?

pour chaque commune, dans chaque école, il faut que l'éducation nationale communique aux maires gestionnaires le nombre de salles où se dérouleront l'enseignement ou d'autres activités,

en insistant sur l'absolue nécessité d'un strict respect du cadre actuellement fixé, et ce jusqu'au 11 mai, et sur l'application, tout aussi stricte, après cette date, d'un ensemble de gestes barrières qui appellent à la responsabilité et au civisme de chacun. Le groupe du RDSE partage globalement le plan présenté : il correspond à une analyse lucide, nourrie d'avis scientifiques, sur l'extrême gravité de cette crise unique dans notre histoire. Nous saluons la volonté de l'État de s'appuyer sur les collectivités territoriales pour la mise en oeuvre de ce plan, en reconnaissant la diversité des situations. Il est bien trop tôt pour tirer des enseignements définitifs de la période que nous vivons, mais probablement arriverons-nous à la conclusion que nous ne sommes efficaces que lorsque les deux puissances publiques que sont l'État et les collectivités se coordonnent parfaitement. Certains

Un collégien prenant les transports publics pourrait avoir besoin de quatre masques pour une journée complète, ce qui se traduirait pour une famille, en prenant en compte les masques des parents, de plusieurs dizaines d'euros par mois, et ce pendant potentiellement de nombreux mois. Si nous avons bien compris que les centres communaux d'action sociale, les CCAS, et les associations pourraient intervenir pour les personnes en situation de précarité, l'État a-t-il prévu une aide pour les ménages salariés modestes pour lesquels cet achat représentera une charge importante et qui risqueraient alors d'utiliser des masques périmés ou ne répondant pas aux normes ? Cette aide pourrait par exemple prendre la forme d'une réévaluation de la prime d'activité et, ainsi, être facilement distribuée par les caisses d'allocations familiales. La parole est à M. le Premier ministre.

précisions.Comme disait l'autre, ce n'est pas votre question, mais c'est tout de même ma réponse ! Vous avez un célèbre prédécesseur, monsieur le Premier ministre ! J'en ai beaucoup, monsieur le président

pour aider à fournir l'ensemble de notre population à compter du 11 mai prochain, j'ai indiqué hier que, pour encourager cette acquisition générale, dès lors que nous avions la certitude que nous pouvions équiper les soignants dans la durée, l'État s'engageait à accompagner

je crois plus juste d'étendre à toutes les commandes de masques passées depuis que le Président de la République a évoqué la date du 11 mai,

et en porter la responsabilité, pour autant, l'état d'urgence sanitaire peut-il justifier un confinement de la démocratie ? Dès le 20 mars, nous avons exprimé nos plus vives réserves sur le transfert massif des prérogatives du Parlement à l'exécutif. Notre inquiétude était malheureusement fondée : depuis cette date, le Parlement est réduit au rôle de figurant. De visioconférence en visioconférence, notre pouvoir de contrôle est mis en scène pour tenter de masquer la réalité : le Président a décidé, le Parlement est écarté du débat.

et moi-même vous demandons, monsieur le Premier ministre, de rendre le pouvoir au Parlement. L'épisode d'hier à l'Assemblée nationale n'est pas acceptable. La mission de la représentation nationale n'est pas seulement de formuler un accord ou un désaccord avec le Gouvernement, sauf à poser la question de confiance.

Le Gouvernement ne serait pas présent quand les parlementaires lui posent des questions ; il ne répondrait pas présent lorsque les commissions permanentes de l'Assemblée nationale ou du Sénat lui demandent de venir leur expliquer ou cela, de travailler et d'exposer des hypothèses qui, parfois, ne sont pas retenues. Le Premier ministre et les membres du Gouvernement ne répondraient pas aux demandes des missions d'information constituées dans telle ou telle assemblée. La vérité, monsieur le sénateur, c'est que, depuis le début de cette crise sanitaire, le Gouvernement a répondu à toutes les demandes formulées par le Sénat

Nous ne vivons pas des temps normaux, monsieur le sénateur. Si l'on pense que l'arsenal juridique préexistant aurait permis de régler la question de l'état d'urgence sanitaire, il faut le dire.

de m'exprimer à l'Assemblée nationale, parce que celle-ci, comme le Sénat, bien entendu, est le lieu où l'on débat des sujets d'intérêt national, le lieu où l'on peut prendre une position. Je l'ai déjà indiqué hier, monsieur le sénateur : les parlementaires ne sont pas des commentateurs de l'action publique ; ils prennent une position politique.

Monsieur le Premier ministre, hier, lors de votre déclaration devant l'Assemblée nationale, vous avez esquissé les conditions du déconfinement scolaire, question qui est évidemment au coeur des préoccupations des familles.

Tout au plus me permettrai-je d'attirer votre attention sur certaines questions qui restent en suspens et méritent, à mon sens, des éclaircissements. D'abord, comment concilier l'urgence pédagogique vis-à-vis des décrocheurs avec un retour en classe basé sur le volontariat ? Ensuite, alors que nos professeurs sont très largement mobilisés, comment assurer à la fois leur présence en cours et le prolongement d'un enseignement à distance pour ceux qui n'auront pas repris le chemin de l'école sur la base du volontariat ? Par ailleurs, il demeure des questions qui concernent directement les compétences des collectivités locales ; elles méritent d'être éclaircies, car beaucoup d'élus nous interrogent. Quelles sont les préconisations du Gouvernement concernant la restauration et les transports scolaires, ainsi que les activités périscolaires ? Qui fournira les masques et qui les paiera ? Toutes ces questions sont importantes. Il ne faudrait pas faire peser sur les épaules des seuls maires la charge de la gestion de cette crise. Je suis convaincu, comme nombre de mes collègues, que les maires mettront que les maires mettront tout en oeuvre pour réussir ce déconfinement, mais ils ne peuvent pas être tenus responsables d'éventuelles contaminations qui auraient lieu au sein des établissements scolaires. Sur ce dernier point en particulier, monsieur le Premier ministre, pouvez-vous leur apporter une garantie ? La parole

la gestion de la crise sanitaire et de ses conséquences, tant sociales qu'économiques, met en lumière le rôle primordial des collectivités territoriales et des élus locaux. Je salue l'engagement de ces femmes et ces hommes et les remercie de l'action menée au quotidien au service de leur population. Tandis que l'État peine à arrêter des orientations claires et à fournir des tests à la population, des masques et équipements aux personnels mobilisés, ce sont les collectivités territoriales qui pallient les manques et, ainsi, assurent la continuité des services, la continuité de l'État. Hier, le Premier ministre a reconnu le rôle essentiel joué par les élus locaux dans cette crise ; ce matin, il a rencontré les associations d'élus dans un exercice étrange : une concertation sur des décisions

Or cette crise pèse lourdement sur les finances des collectivités territoriales. De fait, en métropole comme dans les territoires ultramarins, le confinement a provoqué un effondrement des recettes,

nationale de notre ami Jean-Marie Bockel, pour évaluer la situation des collectivités territoriales. C'est tous ensemble que nous apporterons une réponse

déjà affaiblie par le Brexit avant l'éclatement de la crise sanitaire, peut-elle être aujourd'hui une victime collatérale du Covid-19 ? Alors que nous avons plus que jamais besoin de l'Union européenne, les problèmes européens semblent devant nous intransigeance des pays du Nord à l'égard d'une solidarité européenne plus intégrée, choix américain des Allemands pour l'application de qui laisse la France bien seule sur la scène européenne avec son StopCovid, fermeture des frontières, restrictions de circulation pour les biens et les personnes

comme me l'ont indiqué Claude Kern et mes autres collègues frontaliers, de nombreux points de passage vers l'Allemagne ont été fermés. Les Alsaciens travaillant en Allemagne doivent ainsi attendre des heures aux postes frontières pour des contrôles administratifs et policiers tatillons, une situation qui entraîne des tensions de part et d'autre de la frontière.

pour faciliter la situation des travailleurs frontaliers ? Plus globalement, quels échanges avez-vous engagés avec l'ensemble de nos voisins pour anticiper la sortie de crise et permettre un retour progressif à la normale ?

Létard, nos concitoyens des territoires frontaliers ne seront pas les oubliés du déconfinement. La frontière, qui était pour eux invisible, est subitement réapparue avec cette crise. Je sais le désarroi et la souffrance que cette